Dans l’exercice de territorialisation, les Scot doivent déjà tenir compte de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier.

L’article 3, dans la rédaction issue des travaux de la commission, vise à repousser les délais de modification des documents régionaux de planification et des documents d’urbanisme au minimum nécessaire, afin qu’il puisse être tiré parti des souplesses

il faudrait attendre que les documents soient modifiés avant que ne débute la période de référence. Êtes vous prêts à repousser la période 2021 2031 à 2028 2038 ? Par ailleurs, il ne s’agit ici que d’une date butoir. Rien n’empêche les collectivités qui le souhaiteraient, et seraient prêtes à le faire, de procéder aux modifications dès maintenant.

trop juste pour la collectivité de Corse, ainsi que pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, au regard des contraintes spécifiques liées à la procédure d’évolution de leurs schémas respectifs.

proposition de loi repousse, pour la troisième fois en quatre ans, la date limite de modification des documents régionaux de planification. Il est à présent nécessaire que toutes les régions se mettent en ordre de marche, y compris la Corse

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les collectivités d’ouvrir à l’urbanisation, au travers de leurs documents d’urbanisme modifiés pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des surfaces dépassant de 20 % leur enveloppe foncière théorique, ainsi qu’il en résulte de la déclinaison et de la territorialisation des objectifs fixés dans les documents régionaux de planification. Il s’agit de sécuriser juridiquement

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les surfaces ouvertes à l’urbanisation soient inférieures à l’enveloppe foncière théorique, comme le permet, du reste, le droit en vigueur. Quel est l’avis

Je rappelle, tout d’abord, que je suis défavorable à l’ensemble de l’article 3, sur lequel le Gouvernement a déposé un amendement de suppression. Je partage votre volonté de donner de la souplesse à l’ensemble des collectivités locales dans le cadre de l’aménagement du territoire. Mais, dans la pratique, cet objectif est déjà en partie satisfait

Repousser les délais limites de modification des documents d’urbanisme à 2036 n’est pas cohérent avec l’élaboration d’une trajectoire crédible de réduction de la consommation d’Enaf

M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Pene ; d’autre part, par corrélation, la prohibition des exemptions sectorielles, à l’exception de l’industrie pour laquelle le Gouvernement propose un forfait national exceptionnel, au travers d’un amendement dédié. La réindustrialisation de notre pays est une priorité nationale. Je souhaite donc prendre en compte les besoins particuliers des territoires qui accueillent les projets économiques indispensables au développement

Ainsi, à compter de la date de promulgation de la présente loi, les projets industriels auront vocation à émarger prioritairement sur cette enveloppe, plutôt que sur l’enveloppe des Pene. Cette réserve consiste en un forfait de 10 000 hectares qui sera décompté nationalement, et non dans la consommation des collectivités d’implantation, et qui sera – c’est en cela qu’il est intéressant – mutualisé entre les régions. L’inscription des projets dans l’enveloppe nationale dédiée à l’industrie se fera donc selon une procédure simple, concomitante aux dépôts des autorisations d’urbanisme. Cette procédure, distincte de celle de l’inscription sur la liste des Pene, sera précisée par décret en Conseil d’État. La liste de ces projets sera ainsi rendue publique. Il convient néanmoins de limiter ce mécanisme à ce seul secteur stratégique, le principe de territorialisation devant être l’outil d’absorption des autres secteurs d’activité, hors industrie. Je vous remercie destiné aux projets industriels, afin qu’il atteigne dix ans. Ce prolongement permettrait d’aligner ce mécanisme sur les nouveaux objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d’Enaf définis dans les documents régionaux pour la période 2024 2034, et garantirait ainsi une cohérence stratégique sur le long terme.

Je souhaite prendre en compte les besoins particuliers des territoires ; voilà pourquoi j’ai proposé de substituer aux mesures d’exemption de l’article 4, tel qu’amendé par la commission, un dispositif dédié à ces implantations.

Il est défendu,

n° 49 rectifié. Cet amendement vise à exempter les installations de traitement de tri et de valorisation des déchets du décompte de la consommation d’Enaf. En adoptant cet amendement, nous permettrions aux collectivités de ne pas avoir à arbitrer entre leurs objectifs d’économie circulaire et de sobriété foncière,

réalisés sur leur territoire par des collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de leur insertion territoriale. En effet, à ce jour, seuls les projets de décarbonation bénéficiant de la qualification de Pene sont décomptés du forfait national dans le cadre des objectifs du ZAN. Il importe d’éviter que les quotas d’artificialisation des collectivités ou de leurs groupements concernés soient pénalisés par des aménagements qui, en réalité, sont rendus nécessaires par la présence de Pene

les routes, les écoles ou encore les logements directement liés à la réalisation de ces projets peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale ou d’intérêt intercommunal. En d’autres termes,

uniquement sur l’enveloppe de l’État. Ainsi, les consommations foncières devront s’inscrire dans la stratégie de sobriété foncière que le texte de la commission a instaurée. Je propose en outre d’instaurer un principe d’interdiction : le surcroît de consommations ne pourra pas être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales

de prendre en compte les aménagements de manière adaptée et proportionnée à ce type de situations exceptionnelles. Le Gouvernement propose un forfait national destiné à répondre aux besoins identifiés dans le cadre de la réindustrialisation,

a pour objet de soustraire les projets industriels du calcul de la réduction de l’artificialisation.

acte l’exclusion et la non mutualisation des projets d’envergure nationale ou européenne, qui représentent actuellement un peu moins de 12 500 hectares, au sein des enveloppes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers fixées aux échelons régional et local. Ainsi, ces dernières ne seraient pas grevées par des projets ne relevant pas de l’initiative de la région ou des collectivités locales. Le présent amendement vise à réorienter ces hectares, désormais disponibles, vers la mise en œuvre d’actions de développement économique dans les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme. Cela permettrait, sans remettre en cause ce dispositif auquel les élus demeurent attachés, d’apporter une réponse aux effets pervers de la mise en œuvre de la garantie de développement communal de 1 hectare, qui a parfois pour conséquence de geler du foncier au détriment des enveloppes disponibles pour les autres collectivités. Ainsi les EPCI regroupant un grand nombre de communes de petite ou très petite taille pourraient ils compenser la « perte » de ces hectares, pourtant nécessaires à leur développement économique. Quel est l’avis de la commission ? Cet amendement

au ZAN en 2050. Cela se matérialise dans un objectif chiffré de réduction de la consommation d’Enaf par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédant la promulgation de la loi

que je partage, elle ne me paraît pas opérationnelle. En effet, il n’est pas possible de fixer un objectif de réduction de consommation pour ce type de projets, alors même qu’au cours de la décennie

dans le temps, il y a urgemment besoin de foncier pour réindustrialiser, construire du logement social et développer nos capacités de production d’énergies renouvelables, il faut garder en tête

de transport d’électricité, bénéficient du même régime d’exemption que ces dernières.

Le choix d’une collectivité d’accueillir ou non une implantation industrielle se fait au moment de l’élaboration des documents d’urbanisme, qui peuvent spécifier des règles particulières pour la localisation et la forme de ces implantations. Ce sont ces règles, et uniquement ces règles,

l’ensemble des installations, équipements et infrastructures liés à la production d’hydrogène renouvelable et bas carbone

Dans un souci de cohérence et d’efficacité, les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques doivent bénéficier du même régime d’exemption temporaire que les projets industriels et les projets d’installation de production d’énergies renouvelables auxquels ils sont liés.

Cet amendement vise à donner de la souplesse aux EPCI compétents dans l’aménagement et la gestion des zones d’activité économique (ZAE). Le nombre de ZAE en France est estimé entre 24 000 et 32 000, soit 26 % des surfaces artificialisées.

Autoriser le regroupement d’entreprises liées permettrait aussi de répondre aux enjeux climatiques et économiques, en adoptant des pratiques d’aménagement durables et des logiques de mutualisation et de circularité des ressources.

Il n’est pas réaliste d’exclure du décompte d’artificialisation des sols l’ensemble des infrastructures et constructions qui sont utiles, car beaucoup d’aménagements sont utiles, voire très utiles ! Aussi, même si la prévention du risque inondation est bien entendu un enjeu crucial – je l’ai bien vu dans le département dont je suis élue –, je ne suis pas favorable à ces amendements.

en ce qui concerne le risque inondation, une grande partie de la solution passe par la non artificialisation, voire la désartificialisation. Il y aurait donc un paradoxe à exempter du décompte ces ouvrages et infrastructures. Je demande le retrait de ces deux amendements. À défaut,

Dans les prochaines années, de nouvelles installations seront nécessaires pour assurer une distribution effective à l’ensemble des usagers, mais aussi pour respecter les impératifs de dépollution des eaux destinées à la consommation humaine.

Seule la préservation d’une logique de mutualisation nous permettra d’atteindre l’objectif programmatique national et la rationalisation de l’usage des espaces naturels, agricoles et forestiers.

il n’est pas acquis que les opérations visées par votre amendement emportent systématiquement de la consommation d’Enaf au sens de la loi. Prenons l’exemple des réseaux enterrés : ils ne supposent pas,, de consommation d’espace,

et de l’enseignement technique dans la liste des projets d’envergure régionale, compte tenu de leur intérêt structurant pour les territoires.

par rapport au droit actuel pour adapter les enveloppes aux besoins.

entraîne, à terme, la destruction du bâti patrimonial non protégé, qui se voit progressivement remplacer par des constructions neuves, et ce au détriment de la réhabilitation du bâti ancien, aujourd’hui injustement classé dans la catégorie des passoires thermiques.

dans la circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols », qui permettait déjà de sécuriser juridiquement les collectivités. circulaire, que, « pour une opération d’aménagement prévue en tout ou partie sur des Enaf, l’élément déclencheur de la comptabilisation de la consommation d’espaces n’est pas l’acte administratif de création ou de réalisation d’une ZAC, mais le démarrage effectif des travaux

En effet, la loi Climat et Résilience prévoit d’imputer l’artificialisation résultant d’un projet à la période décennale durant laquelle celui ci sortira de terre, ce qui peut être particulièrement problématique pour les maîtres d’ouvrage d’infrastructures linéaires, de telles opérations ayant

de la conférence régionale de gouvernance de la sobriété foncière. Leur présence

de la territorialisation des enveloppes foncières dans le périmètre régional. Nous avons de plus permis à ces conférences d’enjoindre aux régions de rouvrir le volet artificialisation du Sraddet.

dans le fascicule du Sraddet. Nous observons aujourd’hui que les autres règles relatives à la sobriété foncière figurant dans le fascicule continuent de s’appliquer de manière très contraignante pour les collectivités.

Jean Claude Anglars. La loi impose à la conférence régionale de gouvernance de représenter équitablement les différents types de territoires – urbains, ruraux, de montagne et de littoral.

objectif permet en effet de mieux distinguer les communes peu denses et très peu denses, et d’assurer une représentation cohérente de chaque catégorie de territoire. Pour les communes de montagne et du littoral, je propose un renvoi aux dispositions spécifiques déjà prévues dans la loi. Quel est l’avis de la commission ? Je comprends

L’article 6 de la proposition de loi étend en effet la possibilité, pour une commune, de mutualiser la garantie communale avec une autre commune, à l’échelle du Scot ou à l’échelle régionale.

rendent l’existence de cette garantie plus soutenable pour tous les territoires. Il nous semble logique de maintenir le droit au projet pour les communes rurales, y compris après 2031 ou 2034.

dans les territoires ruraux. Le présent amendement vise donc à protéger spécifiquement les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille de densité communale. Il s’agit de revenir aux dispositions votées par le législateur en 2023 pour éviter que le juge administratif puisse en dénaturer la portée. Quel

Toutefois, la garantie de développement communal permet bien de garantir à chaque commune une enveloppe foncière minimale, qui ne peut pas être réduite au motif d’une absence de croissance démographique ou de dynamisme

c’est la définition de zones à urbaniser au cours de l’élaboration ou la modification du document d’urbanisme qui permet de transcrire concrètement l’existence de la garantie. Je vous demande donc de retirer votre amendement. Quel

au moins un hectare urbanisable dans le PLUi. La mutualisation de cette garantie à l’échelle intercommunale respecte la logique des bassins de vie, consolide la solidarité de proximité et s’intègre dans une dynamique d’aménagement cohérente. En revanche, une mutualisation à l’échelle régionale modifierait profondément la philosophie initiale de cette garantie. Elle risquerait de concentrer les potentiels de développement dans des zones déjà denses en négligeant les spécificités rurales. Les débats parlementaires sur la loi Climat et Résilience avaient bien souligné qu’une telle régionalisation éloignerait les décisions du terrain et aboutirait à une gestion trop centralisée des enveloppes foncières, pénalisant les territoires les moins urbanisés. Cet amendement vise donc à empêcher ce glissement en maintenant l’échelle intercommunale comme le cadre pertinent de la mutualisation. Ainsi, chaque commune conserverait une capacité de développement adaptée à ses besoins réels, en cohérence avec la solidarité territoriale.

Il est difficile de repérer précisément les quelques parcelles qui accueilleront le nouveau projet, d’où la nécessité de multiples révisions. Par cet amendement, je propose donc d’introduire de la souplesse en autorisant, dans la continuité des parties déjà urbanisées, la définition d’un zonage élargi dans lequel le projet pourra s’implanter sous réserve, bien entendu, de respecter la surface maximale permise. Le décompte s’effectuera au moment des autorisations d’urbanisme, permettant une extension urbaine mesurée en adéquation avec la sobriété foncière. Cette souplesse maintient un cap d’urbanisation contrôlée tout en évitant des révisions successives des PLU pour des territoires qui accueillent peu de permis de construire. Elle s’aligne sur l’esprit du RNU et préserve la logique d’un développement progressif, évitant de figer prématurément des parcelles dans un zonage rigide. à l’objet de cet amendement la définition de zones à urbaniser lors de l’élaboration ou de la modification du document d’urbanisme qui permet de transcrire concrètement l’existence de la garantie. Le choix de la localisation des zones à ouvrir à l’urbanisation relève des communes, il n’y a pas de raison de leur ôter cette latitude, uniquement pour mobiliser la garantie de développement communal. L’avis de

Le principe de la garantie de développement communal répond à une volonté partagée de protéger les petites communes dans le processus de territorialisation des objectifs de sobriété foncière.

Voilà